Depuis lors, comme vous le savez, l'assiette du CIR a été étendue au volume total des dépenses de recherche, et le taux majoré a été supprimé. Ainsi cette dépense fiscale a-t-elle atteint 6 milliards d'euros.

À tout le moins, il serait raisonnable de dresser un bilan objectif et chiffré des effets réels du CIR sur la recherche française, avant d'en accroître encore la charge

madame la secrétaire d'État, chers collègues, les effets de la crise de 2008 se sont fait durement sentir outre-mer, où ils ont renforcé la prise de conscience suivante : le moment est venu de trouver les moyens de sortir, par le haut, d'une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance. Dans ce cadre, il est indispensable de favoriser l'implication des grandes entreprises nationales de recherche et de développement. Ces dernières trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens outre-mer. Elles participeraient ainsi à la création d'une masse critique nécessaire

Un levier puissant de cette implantation d'antennes nationales pourrait être l'aménagement du CIR. Pour l'heure, jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses par entreprise ou groupe d'entreprises consolidées, la recherche bénéficie d'un crédit d'impôt de 30 % de la base éligible. Au-delà de 100 millions d'euros, ce crédit d'impôt est réduit à 5 %.

Dans ce contexte, la commission susvisée a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au CIR. Cette

Actuellement, aux termes de l'article 244 B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Le présent amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.

Le scrutin est ouvert.

n° II-2 rectifié . L'engagement des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd'hui freiné par le fait que celle-ci implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l'entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Afin de compenser ces handicaps et d'accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l'environnement et de la biodiversité, cet amendement tend à accorder le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 L du aux exploitants qui obtiennent une certification ouvrant droit à la qualification haute valeur environnementale, ou qualification HVE, en application des dispositions de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime., maritime., le bénéfice de ce crédit d'impôt pourrait être accordé au titre de l'année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée, jusqu'au 31 décembre 2020.

Car c'est un engagement fort qu'a pris la profession viticole depuis ce jour d'avril 2016 où mon collègue Bernard Farges, alors président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, a annoncé la volonté de la filière de sortir progressivement des pesticides. Cette annonce émanant d'un département que je connais bien, la Gironde, a eu l'effet d'une petite bombe. Il est donc indispensable de soutenir la profession dans une démarche qui a vocation à montrer la voie à suivre dans notre pays. Le « tout bio » n'est pas la solution ultime ; d'autres certifications existent. Cet amendement vise à inciter les viticulteurs à s'engager dans une démarche de certification haute valeur environnementale.

aux exploitants qui auraient obtenu une certification ouvrant droit à la qualification haute valeur environnementale. Évidemment, je parle ici d'une certification environnementale de niveau 3, fondée sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, à la stratégie phytosanitaire, ainsi qu'à la gestion de la fertilisation et de l'irrigation. La viticulture consomme peu de pesticides, mais elle en consomme encore 20 %. Il est par conséquent de santé publique d'aider la profession à poursuivre la profonde mutation qu'elle a

évaluation nous sera extrêmement utile pour éclairer le Parlement avant le prochain débat budgétaire.

depuis très longtemps, mais on n'a toujours pas trouvé les dispositifs nécessaires. Or ce sujet est d'une importance majeure pour nos agriculteurs. Dans un contexte de plus en plus imprévisible, l'agriculture n'est pas épargnée par les aléas de toute sorte. Ces facteurs peuvent faire de un à quatre le résultat d'une exploitation et fragiliser à long terme la pérennité des exploitations. Complémentaire à l'assurance, l'épargne de précaution doit justement permettre à l'exploitant de disposer d'une trésorerie grâce à laquelle, le cas échéant, il pourra affronter les aléas susceptibles d'affecter son exploitation. Concrètement, l'exploitant pourra prélever sur un compte bancaire dédié les liquidités qu'il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui seront nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal

Les politiques publiques sont de plus en plus ambitieuses en matière de gestion du bois et des forêts. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un cadre favorable au développement de cette filière fondé sur des objectifs très volontaires pour mobiliser la ressource d'ici à 2035. Les outils fiscaux doivent donc s'inscrire dans cette perspective. C'est le cas pour le dispositif d'encouragement à l'investissement en forêt, le DEFI, dont l'extinction est prévue le 31 décembre prochain. Cet amendement vise à reconduire ce levier : je le rappelle, il incite les contribuables à concourir à la lutte contre le morcellement de la propriété forestière, au développement des travaux forestiers, ainsi qu'à l'organisation économique du secteur. Il s'agit aussi d'aménager fiscalement les quatre dispositifs d'investissement que sont le « DEFI acquisition », le « DEFI assurance », le « DEFI travaux » et le « DEFI contrat » au travers de la modification des plafonds ou de la conditionnalité. Ce levier pourrait être ainsi plus attractif. Quel

pour les produits phytopharmaceutiques recouvre aujourd'hui exclusivement la liste des produits pouvant être utilisés en agriculture biologique, fixée par le droit de l'Union européenne. À ce titre, le taux réduit s'applique déjà à de nombreux produits de biocontrôle.

bénéficieraient notamment à des personnes sans implication dans l'entreprise agricole, à rebours des dispositifs actuels, qui visent à récompenser l'investissement personnel des bénéficiaires.

telles que les groupements fonciers agricoles et les groupements agricoles fonciers. Enfin, nous sommes surpris que cet amendement

En principe, il est acquis que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s'applique pas aux bâtiments ruraux. Le Conseil d'État a jugé utile de subordonner cette exonération à un usage exclusivement agricole. De son côté, l'administration fiscale, par une interprétation restrictive de la jurisprudence administrative, en a déduit que l'exonération de taxe ne s'appliquait pas lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale.

En se fondant sur cette jurisprudence, l'administration fiscale remet en cause intégralement l'exonération de taxe lorsqu'un exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service commerciales. Ainsi, si un viticulteur possède un pressoir sur lequel il pressure et qu'il le met

taxe pour les bâtiments ou les fractions de bâtiment spécialement aménagés pour les activités non agricoles. Ces approches divergentes créent des difficultés d'interprétation sur le terrain.

l'exonération dont bénéficient les bâtiments agricoles est déjà très dérogatoire au regard du principe d'égalité devant l'impôt ; elle doit donc rester limitée aux agriculteurs et aux activités agricoles. L'appliquer à des exploitations commerciales structurées en vue de traiter la production de tiers irait à l'encontre de ce ciblage. ce ciblage. Par ailleurs, des pertes de recettes importantes pourraient en résulter pour les collectivités territoriales. Le maintien de l'exonération peut être admis même lorsque l'activité de pressurage n'est pas effectuée pour les seules récoltes de l'exploitant, si cela n'excède pas certaines proportions. Cette condition est vérifiée au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, qui a notamment considéré que l'exonération devait être remise en cause lorsque les quantités de raisin achetées auprès de tiers représentent, sur plusieurs années, plus de 20 % de la production de l'exploitation- ce qui laisse tout de même une marge importante. En termes d'interprétation, la qualification en activité agricole est une question qui pourra être abordée dans le contexte des réflexions sur la fiscalité agricole. S'agissant de la qualification des bâtiments

prévoit un rapport que le Gouvernement s'est engagé à remettre au Parlement avant le 1 juillet 2018. Ce rapport permettra d'analyser les modalités d'évaluation des établissements industriels, les différentes requalifications et leur impact.

La réponse de Mme la secrétaire d'État n'apporte absolument aucune précision. La question est extrêmement simple : l'exercice d'une activité annexe fait-il perdre le bénéfice de l'exonération

dans un bâtiment ou au sein d'une exploitation, l'utilisation d'une partie des locaux pour une activité annexe ; dans ce cas, on fait le rapport des surfaces.

par ailleurs à sa charge les dégrèvements liés à l'application du seuil de recouvrement, si bien que les communes ne subissent aucun manque à gagner du fait de son application. Organiser un recouvrement triennal serait très lourd et ne me

les AFP -, créées par la loi du 3 janvier 1972, font partie des outils qui contribuent au maintien du pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où ce mode d'élevage extensif est une activité traditionnelle. Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers qui louent des terrains, en les aménageant le cas échéant, à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant ainsi à leur mise en valeur et à la protection du milieu naturel. Elles permettent notamment, par la réunion d'exploitations, de constituer des unités viables. En plus de l'aménagement pastoral, les AFP peuvent réaliser des équipements forestiers et touristiques, et toute action en faveur du maintien de la vie rurale. Afin d'encourager cette démarche collective sur des territoires fragiles, les parcelles comprises dans le périmètre d'une AFP bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération, mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises, doit s'éteindre en 2017. Au regard des retombées très positives qu'apportent ces associations sur les plans à la fois environnemental et économique, le présent amendement a pour objet de reconduire cette Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Toutefois, ce dispositif représente une contrepartie appréciée, qui permet de favoriser l'action publique en faveur de la dynamisation de ces territoires ruraux de montagne. Quel

tire les conséquences de la réforme des valeurs locatives des commerces de centre-ville en les exonérant de taxe foncière. Cette exonération est censée être compensée par un prélèvement sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. Au-delà d'une perte d'autonomie fiscale pour les collectivités locales, cette mesure risque d'aggraver les inégalités entre ces enseignes et les commerces qui ont déjà subi une hausse de leur taxe foncière à la suite de la révision des valeurs Plus encore, cette exonération pénalisera les surfaces commerciales, généralement plus étendues, vis-à-vis des commerces urbains et des sites de vente en ligne. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

l'amendement n° II-665. L'article 45 exonère de cotisation minimum de CFE les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. nous ne sommes pas opposés à cette mesure qui concerne un million de contribuables, avec un gain moyen pour ces derniers estimé à 85 euros. Pour autant, nous sommes inquiets de l'impact de cet article pour les collectivités territoriales la perte de recettes est en effet compensée un mécanisme de prélèvement sur recettes qui correspondra aux bases perdues multipliées par le taux de CFE appliqué en 2018.

au nom de la commission des finances,

Cette situation tend de plus en plus à réduire sensiblement l'autonomie de gestion des collectivités territoriales. Elle a conduit les élus à pratiquer des arbitrages douloureux, d'autant que les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement n'ont pas contribué à améliorer les choses. Les Les dépenses d'action sociale ou de soutien à la vie associative et culturelle ont été réduites, et c'est surtout la part originale des initiatives locales qui a souffert de cette rigidité. La contribution économique territoriale des entreprises ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle. Quant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'évolution incertaine, elle souffre déjà des effets d'éviction que les entreprises ne manquent pas de faire jouer pour alléger leur facture fiscale. De plus, aucune réponse n'est apportée à la question essentielle de la péréquation des ressources, faute de création d'un nouvel outil approprié, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est qu'une compensation et non une recette nouvelle. À notre sens, une vraie réforme des finances locales ne peut pas se réduire au simple remplacement de la taxe professionnelle, recette relativement dynamique, par une cotisation foncière dont la base est étroite et un complément de taxe sur la valeur ajoutée. La suraccumulation de capital financier, y compris à visée spéculative, fondée sur une préemption constante et permanente des richesses créées par l'activité n'est toujours pas découragée ni prise en compte dans l'assiette fiscale de la contribution économique territoriale. C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la contribution économique territoriale en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Il s'agit, de fait, d'accroître la base imposable de plus de 6 000 milliards d'euros ! Cette proposition que nous défendons depuis un certain temps a d'autant plus de pertinence aujourd'hui qu'il faut donner un vrai sens à la péréquation des ressources fiscales des collectivités locales. L'amendement

est à Mme Brigitte Lherbier. Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la diversité des réalités locales pour revenir à une répartition plus juste du produit des prélèvements sur les paris faits dans les hippodromes. Il existe des situations différentes : certains hippodromes se trouvent sur les territoires de plusieurs communes, d'autres se trouvent en intégralité sur le territoire d'une seule commune. Cet amendement vise à opérer une distinction selon deux cas de figure. Premier cas de figure, l'hippodrome est situé sur le territoire d'une seule commune, qui en est propriétaire et qui contribue aux investissements. Dans ce cas, la part du produit des prélèvements en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule. Deuxième cas de figure, l'hippodrome appartient à une société de courses, qui ne bénéficie d'aucune contribution financière de la part des communes sur le territoire desquelles il est implanté. Il est normal, dans ce cas, que les recettes fiscales en question reviennent à l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel l'hippodrome est ouvert au public. Mon amendement tend à mettre en place une allocation du produit

a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale puis par la commission des finances du Sénat sous la précédente législature. En revanche, il n'avait pas été retenu lors de l'adoption définitive de la loi.

lorsqu'ils ne sont pas exploités commercialement. Un transfert systématique du régime des propriétés bâties vers celui des propriétés non bâties aurait des conséquences non négligeables sur les cotisations, non seulement pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,

La répartition de ces bases d'imposition se fait en application de la jurisprudence du Conseil d'État relative à la notion de disposition d'un bien, la base d'imposition de la société civile de moyens devant comprendre les locaux à usage non privatif des membres- le secrétariat, les salles d'attente communes -et celle des membres devant comprendre les locaux qu'ils utilisent matériellement à titre exclusif pour leur activité, principalement le cabinet pour

En outre, imposer les sociétés civiles de moyens sur l'ensemble des locaux pourrait entraîner une perte de ressources pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, si cette proposition était adoptée, le montant de la cotisation due par la seule société ne serait pas nécessairement égal à la somme

Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, qualifiées d'obsolètes et d'injustes par le Gouvernement. En effet, malgré l'exonération de taxe d'habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. est aussi utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales, par le biais du potentiel fiscal. Avec cet amendement, il s'agit donc de généraliser à l'ensemble des départements l'expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l'administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires à la détermination des nouvelles bases locatives,

pour chaque bien, le loyer perçu au 1 janvier 2018. Pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s'inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l'impôt sur les revenus de 2017. Par rapport à l'expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé, comme le conclut le rapport précité. La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision. À l'issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l'année 2019 sur les conséquences de la réforme du point de vue, tout à la fois, des contribuables et des collectivités territoriales. Faute de données relatives à l'ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n'a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales : modification du potentiel fiscal, en particulier, et conséquences sur les dotations et la péréquation. En 2019, le Parlement pourra ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie, mais aussi le calendrier d'entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d'atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable cette réforme.

du Gouvernement ? Les services de mon ministère ne portent pas la même appréciation que la commission des finances du Sénat sur la simplicité ou la lourdeur de la mise en oeuvre de cette expérimentation, que l'amendement tend à étendre à l'ensemble du territoire en 2018.

avait été votée en 2013, a permis d'appréhender la complexité de la démarche. Elle apporte aussi un éclairage fort utile sur l'impact de la réforme. Réaliser une expérimentation nationale en 2018

Le Président de la République a annoncé un chantier plus vaste et plus structurant de refonte globale de la fiscalité locale. Je reconnais bien volontiers que notre système de valeurs locatives est obsolète et injuste, et que la réforme de la taxe d'habitation ne conclut pas ce débat, puisque la taxe foncière sur les propriétés bâties est aussi concernée. Une mission a été confiée à MM. Dominique Bur et Alain Richard sur ces sujets et le Comité des finances locales travaille également sur des pistes de réforme. Il paraît prématuré d'anticiper les conclusions de ces travaux, en lançant dès maintenant une généralisation de l'expérimentation.

les annexes 2042 et 2044 de la déclaration d'impôt sur le revenu, qui sont souscrites par voie dématérialisée. Il suffit que ces annexes soient renseignées

pourrait freiner le marché de l'immobilier et favoriserait les communes dans lesquelles le marché de l'immobilier est dynamique, ce qui déséquilibrerait la répartition des recettes des collectivités territoriales. Pour ces raisons, nous demandons le retrait de cet

est tout à fait compréhensible, elle ne correspond sans doute pas au stade de réflexion où nous sommes. La lettre de mission que M. Dominique Bur et moi-même avons reçue du Premier ministre prévoit bien- j'y avais veillé -que la mise en route de la révision générale des bases locatives

de gestion des déchets. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal apparaît aujourd'hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines, privant ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe. Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collecte de déchets, qui sont éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes.

plutôt que les seules dépenses du service de collecte et de traitement. Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l'annexe relative à la TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets. De plus, l'adoption de cet amendement ne créerait aucun effet d'aubaine.

ont la possibilité de lever une taxe dédiée, en respectant la date d'institution prévue par l'article 1530 du code général des impôts. Selon cet article, ces délibérations devaient être prises avant le 1 octobre 2017. Or cette procédure est parfaitement illégale, puisque les collectivités ne peuvent pas lever une taxe, alors même qu'elles n'ont pas la compétence. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à leur laisser la possibilité

alors que nous ne sommes plus ni présidents de communauté de communes ou d'agglomération ni maires. J'insiste sur l'extrême légèreté avec laquelle ont été traités les communes et les EPCI dans le cadre de cette ineffable loi MAPTAM dont nous subissons encore les conséquences.

de manière marginale le déficit de l'État- j'espère que vous apprécierez -en procédant au relèvement du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale au titre de la valeur ajoutée. La situation est connue : la réforme de la taxe professionnelle a pu s'imposer au motif, entre autres, qu'une part importante de la facture était, en dernier ressort, payée par l'État. Or la naissance de la nouvelle contribution économique territoriale a conduit à la baisse du produit fiscal perçu et, par voie de conséquence, c'est le budget de l'État qui a été le plus avantagé. Mais la combinaison de la CFE et de la CVAE a conduit, peu à peu, à la progression du produit fiscal perçu, et le plafonnement de la valeur ajoutée a recommencé à faire son apparition il n'a pas la même importance que dans le passé, mais il s'agit pour nous d'en éviter une croissance trop rapide. Tel est le sens de cet amendement, qui ramène le taux de valeur ajoutée à partir duquel s'applique le plafonnement à 3,5

et vise à cofinancer des projets concernant les espaces mutualisés de services au public, la rénovation thermique et la transition énergétique, ou l'accessibilité des établissements recevant du public. Pour autant, une interprétation un peu stricte et réglementaire de cet article exclut de l'éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d'équipements publics d'une opération d'aménagement. Dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d'inscrire l'investissement dans son propre budget. L'inscription dans le programme des équipements publics permet d'assurer la réalisation et le financement d'un équipement public dans le cadre d'une opération d'ensemble. De plus, en tant que bien de retour, l'équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession. Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l'article L. 2334-33 du code et à permettre le financement d'équipements publics d'intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d'une concession d'aménagement confiée à une société publique locale, une SPL. Quel est l'avis de la commission

Cet élargissement est assez significatif, puisque le champ d'intervention des SPL est souvent très large et porte sur plusieurs opérations, alors que la DETR vise à soutenir les opérations jugées prioritaires par le Gouvernement. il n'est pas certain qu'un financement des SPL par la DETR soit judicieux juridiquement. L'Autorité de la concurrence a rappelé les conditions très précises à remplir quant au financement des SPL pour assurer sa compatibilité avec le droit communautaire des aides d'État. Ce type de financement nous semble risqué à cet égard. En

Il concerne la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité, afin que le produit recouvré soit reversé aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur leur territoire. Cet amendement est logique, puisqu'il s'inscrit dans une démarche de fléchage des ressources au profit des structures dédiées. Il est tout naturel que des syndicats d'électrification perçoivent le produit de cette taxe ; cela n'a malheureusement pas toujours été le cas dans trop de départements, où elle se trouvait noyée dans les ressources fiscales de toute nature et injectée pour le financement des dépenses de fonctionnement.

aux droits et obligations de l'actuelle collectivité territoriale de Corse et des deux départements : elle percevra la taxe sur la consommation finale d'électricité.

Relations avec les collectivités territoriales ». Notre assemblée, à l'article 60 du projet de loi de finances, a prorogé les incitations financières pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création est compris entre le 2 janvier 2017 et le 1 janvier 2019. Pour les communes nouvelles de moins de 15 000 habitants, cet article prévoit notamment le maintien de la dotation forfaitaire de la DGF au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes, ou encore le versement d'une bonification de 5 % de leur dotation forfaitaire. Les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres

Le succès des communes nouvelles n'est plus à démontrer. Il est largement dû à la loi du 16 mars 2015 qui en a réformé le régime pour le rendre plus souple et plus attractif sur le plan institutionnel et financier, tout en préservant l'identité des communes fusionnées, et surtout en maintenant le caractère volontaire de ces fusions. Or, en l'état actuel, ces incitations se font par un prélèvement sur l'enveloppe DGF, laquelle est fixe et déterminée chaque année en loi de finances. En d'autres termes, les bonifications pour les communes nouvelles se font en diminuant d'autant le montant de la DGF de toutes les autres communes. Le présent amendement vise donc à créer un fonds spécifique dont les ressources seraient prélevées sur les recettes de l'État et qui serait distinct de l'enveloppe DGF. C'est sur ce fonds que seraient financées les incitations pour les créations et les extensions de communes nouvelles.

par rapport au montant total de la DGF du bloc communal. En 2016, par exemple, ces montants se sont élevés à environ 19 millions d'euros, soit 0,1 % de la DGF du bloc communal. Du point de vue des principes, il nous semble justifié que ces garanties

à Mme Jacky Deromedi. Cet amendement prévoit d'élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d'une exonération, en tout ou partie, de la taxe d'aménagement. L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d'aménagement. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d'ouvrage, excluant par là même celles dont le portage est privé ou qui sont initiées par d'autres niveaux de collectivité locale que la commune. Or, face à l'aggravation des déserts médicaux, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière. Aussi, cet amendement prévoit d'étendre cette possibilité d'exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d'initiative publique autre que communale.

Mme Nathalie Delattre. La loi de finances pour 2013 a mis en place un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Pour bénéficier de ce fonds de soutien, les collectivités et établissements concernés avaient jusqu'au 30 avril 2015 pour déposer une demande d'aide. À la suite de mouvements, de regroupements, de fusions et de transformations de collectivités territoriales, les nouvelles entités héritent d'emprunts structurés et d'instruments financiers souscrits par les entités auxquelles elles se substituent. Ces collectivités ou établissements nouveaux ayant été créés après le 30 avril 2015, elles n'ont logiquement pas pu déposer un dossier de demande d'aide auprès de l'État. Aussi, pour les anciennes entités n'ayant pas sollicité le fonds pour leurs emprunts toxiques, il est proposé par cet amendement que les nouvelles entités bénéficient d'une prolongation de la date de dépôt de demande d'aide jusqu'au 30 juin 2018. Cet amendement n'a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l'État. En effet, il ne modifie ni le montant du plafond du fonds ni sa durée maximale ; mais il permet à de nouvelles collectivités d'y être éligibles.

contraint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, l'amendement n° II-359 vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'impact financier résultant de l'enregistrement des déclarations de changement de prénom

du Sénat sur cette question. Quel est l'avis du Gouvernement ? Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers d'état civil pour l'enregistrement des déclarations de changement de prénom à l'état civil n'ouvre pas droit à compensation,

La séance est suspendue.